À l'issue de sa discussion en première lecture par l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances pour 2020 présentait un déficit budgétaire de 93,4 milliards d'euros ; les amendements adoptés par votre assemblée conduisent à dégrader ce déficit de 3,9 milliards d'euros. Cette évolution de l'équilibre budgétaire résulte pour l'essentiel d'une baisse des recettes fiscales nettes de près de 3 milliards d'euros, d'une hausse des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales de 1,5 milliard d'euros et d'une augmentation des recettes des comptes spéciaux de 700 millions d'euros. En premier lieu, les recettes fiscales nettes, hors prélèvements sur recettes, sont minorées de 3 milliards d'euros. Tout d'abord, les recettes de l'impôt sur le revenu sont diminuées de 700 millions d'euros, compte tenu de l'adoption de l'amendement de la commission des finances qui relève le plafond du quotient familial de 1567 à 1750 euros par demi-part pour l'impôt sur le revenu de 2020. Le montant des droits de mutation à titre gratuit est également minoré de 400 millions d'euros, pour tirer les conséquences de l'adoption de l'amendement de la commission, qui augmente l'abattement fiscal applicable aux donations vers les petits-enfants. En outre, le retour sur la rebudgétisation du compte d'affectation spéciale « Aides à l'acquisition de véhicules propres » prévu en PLF implique une minoration des recettes fiscales de 700 millions d'euros, ce qui est sans effet sur le solde, puisque les recettes des comptes spéciaux sont majorées à due concurrence. Ces modifications d'ampleur mises à part, d'autres amendements ont contribué à dégrader le solde. Ainsi, les recettes de taxe sur la valeur ajoutée sont minorées de 200 millions d'euros, pour tenir compte de l'adoption d'un amendement qui prévoit l'application du taux réduit de TVA à 5,5 % pour les opérations de construction et de rénovation de logements locatifs sociaux.

En second lieu, les prélèvements sur recettes au profit des collectivités sont majorés de 1,5 milliard d'euros. Cette hausse résulte principalement de l'adoption d'un amendement créant un prélèvement sur recettes de l'État, pour un montant de 1,1 milliard d'euros, afin de compenser pour les collectivités la perte de recettes induite par la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social. L'année dernière, lors de l'examen du PLF pour 2019, le chiffrage de certaines mesures avait suscité débat, mais nous maintenons que la création de ce prélèvement sur recettes représente 1,1 milliard d'euros, malgré la mention d'un chiffrage différent dans l'exposé sommaire de l'amendement. Ainsi, l'ensemble des votes intervenus au cours de l'examen du projet de loi de finances par le Sénat conduiraient, en l'état, le déficit budgétaire à se dégrader, pour atteindre 97,3 milliards d'euros.

est évalué par le Gouvernement à 139 millions d'euros ; c'est inexact. Il est en réalité nul, dans la mesure où cet amendement vise uniquement à exclure cette dotation du champ des variables d'ajustement. Le coût de l'amendement n° I-107 sur la compensation des exonérations de taxe

Pour l'amendement n° I-264, qui concerne les FDPTP, le surcoût de 139 millions d'euros indiqué dans notre évaluation correspond à l'annulation des minorations successives depuis 2017, ce qui semble être l'intention de l'auteur de l'exposé des motifs. Toutefois le seul dispositif juridique de l'amendement présente un coût neutre, dans la mesure où il s'agit simplement d'exclure à l'avenir les FDPTP des variables d'ajustement ; il ne revient pas sur les minorations antérieures, malgré l'intention de ses auteurs.

amendement adopté par le Sénat introduit deux modifications du dispositif d'accompagnement financier des régions au titre de la réforme de l'apprentissage. Premièrement, il revient sur la reprise des ressources de 11 millions d'euros pour trois régions présentant des dépenses d'apprentissage supérieures aux ressources affectées à cette compétence. Deuxièmement, il étend la période de référence de calcul du droit à compensation de l'État aux exercices 2018 et 2019, alors que le PLF l'a borné à 2017, afin de retenir un niveau de dépenses d'apprentissage représentatif et équitable. Cette modification a pour conséquence directe de majorer l'accompagnement financier en faveur des régions et représente un surcoût pour l'État de 150 millions d'euros, dès 2020. En effet, l'amendement ne renvoie pas explicitement la majoration de l'effort financier Enfin, l'amendement n° I-746 rectifié revient sur la suppression en 2020 de la fraction de TICPE finançant la prime d'apprentissage versée par les régions. Le montant de cette fraction est stabilisé depuis 2007 à hauteur de 230 millions d'euros

Avant de passer au vote sur l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 2020, je vais donner la parole à ceux de nos collègues qui ont été inscrits par les groupes pour expliquer leur vote. Je rappelle au Sénat que, conformément à l'article 42 de la loi organique relative aux lois de finances du 1 août 2001 et à l'article 47 , alinéa 2, de notre règlement, lorsque le Sénat n'adopte pas la première partie du projet de loi de finances, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, chacun des groupes

CRCE. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, avant de donner la position du groupe CRCE sur la première partie du budget pour 2020 qui ne laisse, vous l'imaginez, aucun doute, je veux dénoncer solennellement les conditions inacceptables d'examen par le Sénat du projet de loi de finances. Ce n'est pas tant le nombre des amendements qui pose le plus grand problème, même si cette inflation devrait nous amener à réfléchir à nos méthodes de travail. Mes chers collègues, avec ce débat, nous venons d'inaugurer la méthode d'examen d'un budget à la découpe. pouvons comprendre l'examen en priorité de certains articles ; mais, quand cette méthode devient systématique, elle met à mal la qualité du travail législatif. Ajoutons à cela le dépôt inopiné de dizaines d'amendements par le Gouvernement, que la commission des finances n'a pas eu le temps d'examiner. Il nous faut dès lors statuer sur le fondement du seul avis du rapporteur général, qui subit, comme nous tous, cette anarchie ! Trop souvent, chacune et chacun d'entre nous a le sentiment que l'organisation des débats de notre assemblée dépend essentiellement de l'agenda des ministres. Enfin, comment accepter cette interruption de nos travaux dimanche matin à zéro heure trente-cinq, quand nous avions collectivement décidé d'examiner les articles jusqu'à trois heures du matin ? Aucune explication officielle ne nous a été fournie à cette Mes chers collègues, il me semblerait salutaire que le Sénat, dans sa grande diversité, exprime sa désapprobation auprès du Gouvernement. Nous avons droit à plus de considération ! Il y va du respect des institutions de la République et de nos concitoyens.

Sur le fond, le Gouvernement a mis en avant la baisse de l'impôt sur le revenu. Bien entendu, la TVA, impôt qui pèse quasiment deux fois plus lourd, 130 milliards d'euros, n'est pas remise en cause de près ou de loin. Sur ce point, la majorité sénatoriale est pleinement d'accord avec le Gouvernement. Notre proposition de réduire la TVA sur les produits de première nécessité et, parallèlement, de la renforcer sur les produits de luxe a été balayée d'un revers de main. Le Gouvernement, bien entendu, a maintenu l'abrogation de l'ISF. il fait fi de l'exigence partagée par une immense majorité de nos concitoyens- plus de 70 % -d'une imposition des grandes fortunes, qui, elles, se portent on ne peut mieux. Nos compatriotes- c'est aussi un constat dans de nombreux pays en ébullition dans le monde -ne supportent plus ces inégalités croissantes, inacceptables, cette concentration de la richesse du monde dans les mains de quelques dizaines d'individus, dirigeants de ces super multinationales qui ont pour objectif ultime, ni plus ni moins, de diriger le monde.

En étranglant financièrement les communes, vous entendez les mettre au pas, les pousser à la contractualisation, qui débouchera fatalement sur la déchéance du service public et la perte d'autonomie financière des collectivités. Sur le plan de l'écologie et de la transition énergétique, qui ont occupé une partie importante de nos débats, comment ne pas constater le décalage entre les intentions affichées et la faiblesse des moyens mobilisés ? Vous l'avez compris, mes chers collègues, mon groupe votera contre cette première partie du PLF pour

Ce budget de mi-mandat doit lancer l'acte II du quinquennat. Comme cela a déjà été souligné lors de la discussion générale, ce PLF pour 2020 s'articule autour de quelques grands axes structurants, tout particulièrement la baisse des prélèvements obligatoires, le verdissement progressif de nos impôts et, bien évidemment, la réforme de la fiscalité locale. Comme nous l'avons rappelé lors de l'ouverture des débats, ce budget présente des avancées significatives sur le plan macroéconomique. Le déficit public est désormais stabilisé sous la barre des 3 % du PIB et le taux des prélèvements obligatoires diminue tant pour les ménages que pour les entreprises. Cependant, la dette continue d'augmenter. Le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat contenait déjà de nombreuses mesures demandées de longue date par notre assemblée. Je pense notamment à celles qui visent à simplifier le maquis des taxes inefficaces, ainsi qu'à la baisse de l'impôt sur le revenu pour les ménages les plus modestes. De même, les dispositions relatives à la fiscalité énergétique seront appliquées de façon plus progressive et moins brutale ; nous pouvons espérer qu'elles recevront un accueil plus chaleureux que celles qui ont Le Sénat a largement amendé le texte, en veillant toujours à préserver les intérêts des collectivités territoriales. Les ajustements apportés aux articles concernant la domiciliation fiscale des dirigeants d'entreprise ou la baisse de l'impôt sur le revenu me semblent ainsi limiter les effets de bord de ces mesures, qui vont dans le bon sens. D'autres dispositions, telles que la redéfinition de l'IFI ou la simplification du régime des donations aux aux petits-enfants, sont la preuve que notre assemblée ne se contente pas du texte qui lui est soumis, mais demeure au contraire force de proposition. Le groupe Les Indépendants a pris sa part à ce travail d'amendement, que ce soit pour ajuster des propositions opérationnelles ou pour lancer des débats de fond. Je pense notamment aux améliorations apportées au régime fiscal des transmissions d'entreprise, ainsi qu'à notre proposition réitérée d'instaurer une TVA sociale, afin de faire basculer les prélèvements obligatoires du travail vers la consommation. Lors de nos débats, c'est tout naturellement sur le volet de la fiscalité locale que l'attention s'est concentrée et que les divergences se sont cristallisées. Mais cette année, ce n'est pas tant le principe de la réforme qui a été discuté porté sur le calendrier d'exécution, donnant lieu à de nombreux débats techniques et à autant d'arbitrages paramétriques, dans un seul objectif : veiller à ce que les collectivités territoriales ne perdent pas au change dans ce grand bouleversement. Le Sénat a donc entériné le report de la réforme. Cette décision me rappelle la fin du roman d'Alexandre Dumas. La chambre haute, tout comme le comte de Monte Cristo, semble convenir que toute la sagesse humaine se trouve dans ces deux mots : attendre et espérer. Attendre de voir quels pourraient être les effets de la réforme de la fiscalité locale avant de la mettre en oeuvre, tout en en acceptant le principe. Espérer que ses résultats ne feront aucun perdant parmi les collectivités territoriales par le jeu des compensations, tout en exhortant l'État à réduire son déficit. C'est sans doute le rôle du Sénat que de faire montre de circonspection et de ne pas céder à la précipitation. Le groupe Les Indépendants partage la volonté de compenser à l'euro près la suppression de la taxe d'habitation pour les communes : cette compensation nous paraît juste et nécessaire. Il veillera à ce que les départements ne se trouvent pas plus mal lotis après la réforme qu'avant. Mais rien ne nous oblige pour autant à repousser cette réforme fiscale, qui a déjà été largement annoncée et qu'une partie non négligeable de l'opinion publique attend. Dans ces conditions, il ne nous semble pas opportun de la renvoyer à un horizon qui, sur le plan politique, paraît bien lointain. Compte tenu de cette réserve importante sur l'approbation de cette réforme, le groupe Les Indépendants s'abstiendra sur le vote de cette première partie du PLF. En tout état de cause, le Parlement continuera à veiller à ce que la compensation, quel que soit le mode de calcul qui sera finalement retenu, préserve effectivement l'autonomie financière de nos collectivités territoriales, singulièrement celle de nos communes. Il y va de la vitalité démocratique de notre pays. Nous veillerons également, lors de l'examen de la deuxième partie du PLF, à ce que les dépenses n'aggravent pas le déficit public. Excellent

Une fois encore, les votes ont transcendé les clivages sur un grand nombre de sujets : imposition des personnes et des sociétés, ressources des collectivités, verdissement de la fiscalité. C'est là la marque de fabrique du Sénat : travail de fond et intérêt général l'emportent sur les postures incantatoires. Cependant, la contrainte d'un calendrier resserré nous a conduits à examiner cette première partie de budget à un rythme effréné, peu compatible avec la clarté du débat démocratique. La difficulté fut par ailleurs renforcée cette année par un ordre d'examen des articles pour le moins dispersé. Je n'y reviens pas. Nous nous réjouissons néanmoins des progrès accomplis en termes d'évaluation de nos décisions. En matière d'impôt sur le revenu, le simulateur LexImpact nous a permis d'être force de proposition et d'animer le débat sur la nécessaire refonte de notre système fiscal. Gageons que cet instrument sera pérennisé et à l'avenir étendu à d'autres impositions que celle des revenus. Au cours de la discussion générale, notre collègue Bernard Delcros vous indiquait que le groupe Union Centriste abordait positivement ce projet de loi de finances. Les débats ont confirmé notre satisfaction sur bon nombre de points. Ainsi en va-t-il de la baisse de 5 milliards d'euros d'impôt sur le revenu au bénéfice des premiers déciles. Nous saluons également la poursuite de la diminution de l'impôt sur les sociétés, dont la trajectoire devra être tenue d'ici à la fin du quinquennat. Nous y veillerons. Les débats ont aussi produit quelques fruits dans le domaine de la fiscalité des donations et des successions. Sur notre initiative et sur celle d'autres groupes, le Sénat a adopté un allégement des droits de mutation à titre gratuit visant à protéger les exploitations viticoles et agricoles familiales. L'enjeu est non seulement le dynamisme économique, mais aussi l'aménagement de nos provinces. Je tiens également à saluer l'abaissement, sur l'initiative du groupe Union Centriste, du délai de rappel fiscal des donations. Il est plus que nécessaire d'adapter notre fiscalité au vieillissement de la population et au déploiement de nouvelles formes de solidarité. J'en viens maintenant au point d'orgue de ce budget pour 2020 : la suppression entérinée de la taxe d'habitation pour 80 % des contribuables et le coup d'envoi de la réforme de la fiscalité locale.

les avancées, je retiens la revalorisation des valeurs locatives dans les conditions du droit en vigueur, c'est-à-dire à hauteur de 1,2 %. Je signale aussi le renforcement du mécanisme de garantie du montant des fractions de TVA affectées aux départements.

tout le monde s'accorde à dire que les comportements doivent évoluer, sans exclusive. En outre- Vincent Delahaye l'a rappelé -, bien d'autres impôts ont une vocation redistributive.

Ce troisième projet de loi de finances du quinquennat s'inscrit parfaitement dans l'orientation libérale du Gouvernement de préservation des intérêts des plus aisés. Certes, sur plus de soixante-dix articles de première partie, nous trouverons toujours des mesures sympathiques ou utiles : c'est indéniable et c'est heureux, aurait dit mon collègue Claude Raynal. Mais la réalité, c'est que ni le Gouvernement ni la majorité sénatoriale ne souhaitent réellement réorienter la politique conduite aujourd'hui dans notre pays : nous ne pouvons que le regretter. La présentation de notre contre-budget démontre qu'une autre politique est possible. Nous avons fait le choix d'axer nos propositions sur trois enjeux que nous jugeons prioritaires : la justice fiscale et sociale, la transition écologique et le renforcement de nos territoires. à l'aune de ces trois priorités, nous ne pouvons qu'être déçus par le volet « recettes », tant dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale que dans la version soumise, en cet instant, au vote de la Haute Assemblée, après être passée au crible de la majorité sénatoriale.

Vous n'avez pas non plus voulu d'un rééquilibrage de l'effort fiscal demandé à nos concitoyens ; vous avez fait le choix de protéger les plus aisés d'entre eux, contre toute logique, si ce n'est idéologique.

Nous vous avons proposé une logique moins coûteuse pour les finances publiques et plus redistributive : vous l'avez rejetée, et notre proposition de rééquilibrage des droits de succession n'a pas connu un sort plus heureux.

Contrairement au Gouvernement, nous croyons en l'intelligence des territoires. Nous nous réjouissons de la position prise par le Sénat, à une très large majorité, concernant la taxe d'habitation. Elle permettra de mieux travailler la problématique de la compensation des collectivités- je pense notamment à l'impact de cette réforme sur

au terme de la première partie du projet de loi de finances pour 2020 et notre marathon fiscal aura été particulièrement dense, avec plus de 1 000 amendements examinés.

partie a été rendue plus ardue par un ordre d'examen des articles quelque peu chaotique. Cette méthode n'a pas toujours favorisé la clarté et la prévisibilité de la discussion, au grand dam de M. le rapporteur général.

Puis, après une séance finalement écourtée samedi soir, nous avons repris hier à un rythme soutenu pour aborder les questions, sensibles, de fiscalité écologique. Se trouve ainsi résumé, en quelques mots, ce que chacun a pu constater, à savoir la complexité du débat budgétaire-

Plus généralement, ce budget se situe exactement à la moitié du quinquennat. De ce fait, il comporte des mesures s'inscrivant dans la continuité des deux lois de finances précédentes. L'article 5 en offre un bon exemple, avec la suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale pour 80 % des ménages, comme annoncé au début du mandat. mandat. La Haute Assemblée a jugé nécessaire de reporter la réforme du financement des collectivités territoriales, trop peu satisfaisante et trop peu lisible. Il est vrai que les transferts et compensations prévus, bien qu'étant à l'euro près, ne sont pas sans susciter des inquiétudes chez les élus locaux, surtout à quelques mois des élections municipales. En revanche, le Sénat a entériné l'abaissement à 11 % de la deuxième tranche d'impôt sur le revenu. Fait intéressant, cette baisse d'impôt s'accompagne en réalité de recettes supplémentaires, qui seraient à mettre au crédit de la réforme du prélèvement à la source. L'impôt sur le revenu et la fiscalité du patrimoine suscitent toujours d'importants débats. Les élus du RDSE sont traditionnellement attachés à l'idée d'impôt citoyen qu'incarnait à l'origine l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, les formes d'imposition sont multiples- impôt sur le revenu, TVA, CSG, CRDS, etc. -et le lien entre impôt et citoyenneté s'est malheureusement abîmé. Par le biais de nos amendements, nous donnons l'alerte et nous tentons de remédier à cette situation, alors que nous constatons, aujourd'hui, une réelle crise du consentement à l'impôt. passe également par une plus grande attention portée à la fiscalité du numérique. Aujourd'hui, des acteurs majeurs de ce secteur peuvent s'acquitter d'impôts très faibles, alors qu'ils dégagent d'importants comporte des mesures permettant de lutter contre l'optimisation et la fraude à la TVA des plateformes, notamment par la transposition de textes européens. Je salue également l'adoption de l'amendement de mon collègue Yvon Collin, tendant à ce que les « pure players » du commerce de détail, c'est-à-dire les entreprises opérant uniquement des commandes en ligne, s'acquittent de la taxe sur les surfaces commerciales. Oui ! Dans le domaine de la fiscalité des entreprises, si les gros acteurs tirent leur épingle du jeu, les petits rencontrent davantage de difficultés, en particulier du fait de la diversité des régimes applicables. l'on peut regretter que n'aient pas été adoptés certains amendements tendant à harmoniser les régimes d'imposition des bénéfices pour les microentreprises, en particulier les micro-exploitations agricoles. Au dossier de la fiscalité énergétique, de nombreuses modifications ont été adoptées, compte tenu de la très grande diversité des activités et des produits concernés. Le Sénat s'est efforcé de préciser le texte, bien que les défis soient immenses. La hausse de la taxe sur les billets d'avion a une forte charge symbolique. Toutefois, cette mesure peut avoir de grandes conséquences dans certains territoires mal desservis. L'amendement de notre collègue Josiane Costes, tendant l'entrée en vigueur de cette hausse sans la supprimer, permettra ainsi de protéger les petites lignes aériennes, indispensables au désenclavement de divers territoires ruraux.

Je mets aux voix, modifié, l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 2020. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit. Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2019

sans obérer le fait que nous n'approuvions pas certains choix, budgétaires et fiscaux, opérés dans le budget initial. Les quatre amendements adoptés tendaient à revenir sur des annulations de crédits que nous avions identifiées

La réussite de la commission mixte paritaire sur ce projet de loi de finances rectificative est donc particulièrement notable, puisque la dernière CMP conclusive en la matière remonte à 2010. que le projet de loi de finances rectificative présenté par le Gouvernement soit modifié sur deux points : le rétablissement de 13 millions d'euros de crédits de la mission « Recherche », d'une part, et le rétablissement de 25 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 21 millions d'euros en crédits de paiement sur le programme « Patrimoines ». Au total, cela représente 38 millions d'euros de moindres annulations en autorisations d'engagement et 34 millions d'euros en crédits de paiement. Le Parlement a donc ainsi exprimé son avis et fait valoir ses positions sur le schéma de fin de gestion proposé dans le Ce PLFR contribue pour partie au financement des mesures d'urgence économiques et sociales, conformément aux annonces du Premier ministre au mois de décembre 2018. Il met en oeuvre cet engagement en dégageant 1 milliard d'euros d'économies sur le champ des dépenses pilotables de l'État de l'exercice 2019. La réussite de cette commission mixte paritaire nous offre l'occasion de saluer la qualité du travail parlementaire pour parvenir à un texte de compromis entre les deux chambres. C'est aussi, ne boudons pas notre plaisir, l'occasion de démontrer que les efforts que nous avons collectivement fournis portent leur fruit. Depuis plus de deux ans,

Nous construisons nos projets de textes financiers sur des hypothèses crédibles et réalistes ; nous procédons à une budgétisation qui tient compte des besoins réels et nous ne recourons plus à aucun décret d'avance, c'est à souligner. Nous avons souhaité et permis que la portée de l'autorisation parlementaire en matière budgétaire soit réellement revalorisée. La réussite de cette commission mixte paritaire montre que nous avons eu raison et qu'il faut continuer dans cette voie. cette voie. Un projet de loi de finances rectificative sans aucune mesure fiscale est une amélioration incontestable pour la clarté des débats, ainsi que pour la prévisibilité de la norme fiscale pour les particuliers et les entreprises. Je me réjouis d'ailleurs que ce point ait été unanimement salué au Sénat et à l'Assemblée nationale. Au-delà de ces avantages qui ont séduit la représentation nationale, c'est grâce à vous, parlementaires, que la méthode proposée par le Gouvernement et qui implique, nous en sommes conscients, des délais contraints d'examen semble validée. Je suis intimement convaincu que l'autorisation parlementaire reprend d'autant mieux sa signification et sa portée que les débats se concentrent sur un nombre raisonnable de dispositions, que le PLFR ne comprend pas de mesures fiscales nouvelles et que l'exécution budgétaire se réalise sans décret d'avance. Je vous remercie d'avoir joué le jeu en ne déposant aucun amendement fiscal. Je forme le voeu que cette méthode prospère et je me réjouis, au nom du Gouvernement, de la réussite de cette commission mixte paritaire.

Ce projet de loi de finances rectificative, quant à lui, souligne l'absence d'ambition du Gouvernement pour nos politiques publiques et pour le mieux-vivre de nos concitoyens.

au lieu de les laisser à disposition pour développer ou rénover des infrastructures, pour créer de nouveaux services, bref, pour améliorer la vie des gens. Le Gouvernement s'est largement félicité de ce collectif budgétaire, constatant en particulier un déficit réduit par rapport aux prévisions de début d'année et un nombre limité d'annulations de crédits.

grâce au durcissement des critères d'attribution consécutif à la réforme du CITE. Conscient de l'impérieuse nécessité d'entamer une transition écologique et de son coût nécessaire,

de nombre de missions, comme je viens de le démontrer. Somme toute, l'amélioration est limitée. Loin de moi l'envie de casser l'enthousiasme du Gouvernement dans sa campagne d'autopromotion,

Pour subventionner la rente de quelques milliardaires, le Gouvernement va davantage creuser le budget de la sécurité sociale et viendra ensuite expliquer aux chômeurs qu'ils ne doivent plus abuser des droits qui leur permettent de vivre entre deux emplois, aux futurs retraités qu'on vit plus longtemps et qu'ils devront donc travailler toujours plus ou vivre dans la pauvreté

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous nous prononçons aujourd'hui sur les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2019, alors même que nous venons tout juste de terminer l'examen de la première partie du projet Voilà qui nous oblige à un troublant exercice d'aller-retour dans le temps. Cette superposition chronologique découle du désaccord survenu à l'issue de la première lecture. de la première lecture. L'Assemblée nationale avait adopté sans modifications le texte du Gouvernement qui ne contenait ni mesure fiscale ni décret d'avance, conformément à la vocation initiale du PLFR.

d'un côté, certains reprochaient au Gouvernement sa prétendue incapacité à réduire la dépense publique et l'exhortaient à toujours plus de sincérité et de rigueur dans l'exécution du budget, de l'autre, on amendait un PLFR qui ne contient pas de mesure politique, pour y supprimer des annulations de crédits, et donc imposer de nouvelles dépenses, tout en saluant la sincérité dans l'exécution du budget. Ce n'est pas facile à comprendre Le groupe Les Indépendants se réjouit, toutefois, que les discussions de la commission mixte paritaire aient pu aboutir et, en particulier, que le point soulevé par le Sénat concernant la mission « Défense » ait été éclairci.

Nous avions déjà soulevé ce point en première lecture. Mon groupe continuera à veiller à ce que nos forces armées, qui sont aujourd'hui confrontées à une période d'instabilité géopolitique inédite, ne pâtissent pas de la volatilité budgétaire qui caractérise notre pays.

liberté. Le même principe guidera l'action du groupe Les Indépendants lors des discussions sur la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2020. Il est toujours facile de prôner dans le discours plus de rigueur sur les grands équilibres et de montrer du doigt quelques grands chiffres, tels que le taux d'endettement ou le déficit public. cependant, lorsqu'il faut décider mission par mission, ligne par ligne, des crédits qui diminueront, lorsqu'il faut assumer d'importantes économies, que les positions politiques se cristallisent. Cette année encore, la ligne de mon groupe sera claire : nous soutiendrons toutes les mesures qui réduisent la dépense publique, sauf celles qui visent l'exercice des missions régaliennes de l'État,

réduit à sa vocation initiale- solder les comptes de l'année qui s'achève -que de redonner du sens à nos débats et de renforcer nos engagements politiques. À quoi bon, sinon, discourir à l'automne sur les crédits de paiement et les autorisations d'engagement de toutes les missions, pour se dédire un an plus tard ? fort, alors, d'affaiblir la voix du Parlement qui autorise l'État à lever l'impôt. C'est pourquoi l'engagement du Gouvernement à présenter chaque année un PLFR

En tout état de cause, le groupe Les Indépendants votera le projet de loi de finances rectificative pour 2019 tel qu'issu des discussions de la commission mixte paritaire.

à ce qui était prévu dans la loi de finances initiale. Nous en sommes heureux pour notre pays et pour nos concitoyens, mais- parce qu'il y a un « mais » -nous n'avons toujours pas réussi à trouver ces recettes supplémentaires. Se

C'est dans cette logique, sans doute, que vous avez choisi, lors de la commission mixte paritaire, de revenir sur ce déblocage de crédits, comme sur d'autres que le Sénat vous avait proposés. Il faut le dire très clairement : nous sommes dubitatifs, pour ne pas dire choqués, par cette décision et par la logique qui la sous-tend. Comme le rapporteur général de l'Assemblée nationale l'a indiqué, les crédits du loto du patrimoine ont été maintenus, sans doute grâce à la pression médiatique de Stéphane Bern. Cela veut-il dire, mes chers collègues, que ce dernier, pour qui j'ai le plus grand respect,

Voulez-vous nous faire croire, monsieur le secrétaire d'État, qu'il n'était pas possible de prendre une décision d'urgence visant ponctuellement à octroyer des fonds supplémentaires aux bénéficiaires des crédits du programme « Vie étudiante », en attendant de pouvoir trouver une solution plus durable ? Là encore, nous aurons la réponse le 5 décembre

La politique, c'est faire des choix, et nous ne pouvons qu'être en désaccord avec les vôtres, qui renforcent les plus forts et fragilisent les plus faibles, non sans un certain cynisme.

Les deux chambres n'ont rien à gagner à s'ignorer l'une l'autre ou à se faire concurrence. Il serait heureux qu'une telle issue soit plus fréquente, sans rien renier des spécificités de chaque assemblée. De façon plus prosaïque, cet accord a le grand mérite de nous faire gagner du temps dans un agenda législatif chargé. Avec ses trois amendements adoptés en première lecture, le Sénat a joué son rôle de contrôle de l'exécution des crédits. Il a été entendu. Nous avons ainsi montré notre vigilance quant au respect de l'autorisation donnée en loi de finances initiale. initiale. Le projet de loi de finances rectificative permet au Parlement d'augmenter les crédits, ou plutôt d'annuler des annulations, sans risquer de tomber sous le coup du redoutable article 40 de la Constitution : la marge de manoeuvre est très faible, mais il a su l'utiliser. L'amélioration du solde, de 10 milliards d'euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2019, est une excellente nouvelle, même si elle est surtout due à la baisse de la charge de la dette par le jeu de taux d'intérêt nuls, voire négatifs, sur lesquels nous n'avons pas prise.

L'évolution des effectifs de la fonction publique d'État aura été nulle en 2019, ce qui marque une inflexion importante par rapport aux annonces du début de mandat, mais à laquelle on pouvait tout à fait s'attendre, compte tenu de la complexité du sujet et des limites d'une approche purement comptable. Plus que par des baisses ou des hausses d'effectifs ou de moyens, trop importants dans certaines administrations, notamment centrales, trop faibles dans d'autres, les politiques publiques passent par une définition claire des missions et des priorités et par une stratégie.

Je constate la hausse des crédits de l'agriculture pour assurer des contrôles sanitaires en vue de l'ineffable Brexit, qui montre que les autorités s'organisent pour affronter les difficultés qu'il pourrait engendrer, quoi qu'il advienne. Je salue le refinancement de 13 millions d'euros de la contribution française à ITER, projet majeur avec lequel se joue une partie de notre avenir énergétique et que nous devons encourager. Les autres mesures d'ouverture ou d'annulation de crédits, la perte de recettes de 400 millions d'euros du compte d'affectation pour les raisons que l'on connaît, celle de 1 milliard d'euros du CAS « Transition énergétique » et, de façon plus générale, la plus grande sincérité budgétaire ont déjà été soulignées en première lecture. L'Assemblée nationale

Encore jeune dans la fonction parlementaire, je découvre les règles qui fixent le calendrier et les modalités d'examen des lois de finances. Le Parlement a besoin de plus de temps, de conditions d'examen plus favorables plus favorables et d'outils d'évaluation plus performants, tant sur les grandes données macroéconomiques que sur l'impact des mesures qu'il propose. Sur le plan du calendrier, je trouve surprenant que le budget de la Nation soit examiné un week-end, ce qui oblige les services à des efforts particuliers- je salue leur engagement pour que notre démocratie puisse s'exercer -et conduit à un examen des amendements, pourtant filtrés avec zèle, dans des conditions peu soutenables. Quoi qu'il en soit, notre tâche est grandement facilitée par la décision du Gouvernement, reconduite cette année, de ne pas présenter d'articles fiscaux dans le projet de loi de finances rectificative. Nous renouons ainsi avec la vocation initiale de ce texte : clore la gestion de l'exercice en cours. En présentant un texte qui respecte ce cadre, le Gouvernement respecte l'autorisation budgétaire donnée dans la loi de finances initiale. Rappelons-nous la pratique passée

de crédits visent aussi à couvrir le dynamisme de la prime à la conversion et du bonus écologique, qui permettent aux Français d'acheter des véhicules propres. Cette tendance montre la volonté des Français d'agir pour la transition écologique.

Une croissance annuelle de 1,3 %, inférieure de 0,1 point à la prévision du projet de loi de finances initial, 97,6 milliards d'euros de déficit budgétaire, contre 96,3 milliards d'euros prévus en septembre dernier,

non ! Certes, les recettes sont révisées à la hausse, de 1,6 milliard d'euros pour l'impôt sur le revenu et de 3,5 milliards d'euros pour l'impôt sur les sociétés, du fait, notamment, de la réforme du prélèvement de l'impôt sur le revenu et de la transformation du CICE en baisse de charges.

ce projet de loi de finances rectificative de fin d'année comportait d'importantes annulations de crédits avant les modifications intervenues en commission mixte paritaire, à hauteur de 1,7 milliard d'euros, hors masse salariale, sur des crédits mis en réserve.

Il faut tout de même rappeler que le Gouvernement n'avait pas jugé utile de justifier cette annulation, portant sur 29,6 millions d'euros en autorisations d'engagement et 25,5 millions d'euros en crédits de paiement, des montants à rapporter à la recette du loto du patrimoine. Remerciez le Sénat, monsieur le secrétaire d'État, d'avoir attiré l'attention de l'Assemblée nationale sur ce point. Je ne crois pas que les millions de Français qui ont joué pour contribuer à la restauration de notre patrimoine auraient apprécié d'être ainsi floués Quant à la mission « Recherche et enseignement supérieur », le Sénat a rétabli 13 millions d'euros qui seront engagés au titre de la contribution française au projet ITER. Il s'agit seulement de permettre à la France de respecter ses engagements internationaux, ce qui relève du bon sens. D'ailleurs, l'Assemblée nationale est convenue du bien-fondé de cet amendement du Sénat.